de la commission des affaires européennes. Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute. Monsieur le ministre délégué, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui ci aura retrouvé

Madame la présidente, madame la vice présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, monsieur le président de la commission des affaires européennes, les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis honoré de me trouver devant vous aujourd’hui afin de vous présenter les principaux sujets qui seront traités lors du Conseil européen des 21 et 22 mars. Je souhaite également profiter de cette occasion pour prendre un peu de recul, sept ans après le discours de la Sorbonne, et alors que, avec les élections européennes, se clôtureront la mandature du Parlement européen et, plus largement, le cycle institutionnel européen. européen. Ce sommet européen se tiendra à un moment charnière pour l’avenir de l’Europe. Ensemble, les chefs d’État et de gouvernement aborderont des sujets prioritaires pour l’Union : le soutien à l’Ukraine, l’Europe de la défense, l’avenir d’une Europe élargie, le conflit au Proche Orient, le soutien à nos agriculteurs, la préparation de l’agenda stratégique, ainsi que la réponse aux défis migratoires. Si l’on s’arrête un instant sur l’ordre du jour de ce Conseil européen, on constate qu’il n’y a pas un sujet qui ne reflète les priorités de l’agenda de souveraineté tel que dessiné par le Président de la République dès 2017, puis décliné à l’occasion du sommet de Versailles, au lendemain du début de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Face aux chocs et aux crises inédites que notre Union a vécus et continue de vivre, le combat que la France a mené dans le but d’arrimer le projet européen à cette ambition a peu à peu résonné chez nos partenaires et trouve plus que jamais un écho en Europe. Très tôt, la France a ainsi appelé de ses vœux une Europe forte dans le monde, capable de parler d’une seule voix et de prendre en main sa sécurité. Nous avons conduit un véritable plaidoyer en faveur d’une plus grande convergence stratégique et de l’avènement d’une Europe de la défense qui assume sa propre sécurité de manière croissante, en complémentarité avec l’Otan. La pandémie et la guerre ont toutes deux joué un rôle de catalyseur vis à vis de la souveraineté européenne. L’invasion russe de l’Ukraine, en particulier, a conduit les États membres à briser ensemble des tabous et à transcender des lignes que nous pensions immuables. Certains de nos partenaires européens nous disent : « Les idées que nous adorions détester il y a encore quelques années sont désormais devenues nos idées ! la Pologne a massivement investi dans ses capacités de défense et le Danemark, à l’issue d’un référendum historique, décidait de rejoindre la politique commune de sécurité et de défense. En quelques jours seulement, nous avons été capables de décider, de façon inédite et historique, de recourir à la Facilité européenne pour la paix (FEP) afin de financer des livraisons d’armes à un pays en guerre. Aujourd’hui, face à une Russie qui mise sur l’incapacité des partenaires de l’Ukraine à la soutenir dans une guerre longue, il nous faut poursuivre nos efforts et approfondir la réflexion sur les modalités de notre soutien, sans tabou, pour faire plus, mieux et différemment, à l’instar de l’initiative engagée par le Président de la République le 26 février dernier. est bien l’esprit du sommet de Versailles, lequel, quelques semaines seulement après le retour de la guerre sur le continent européen, avait contribué tout à la fois à concrétiser le réveil stratégique européen et à poser les premiers jalons d’une base économique et industrielle européenne plus solide, tournée vers le renforcement de ses capacités de production. Tirant également les leçons de la pandémie de covid 19, l’agenda de Versailles avait constitué un tournant essentiel pour l’Europe en visant la réduction de nos vulnérabilités et dépendances stratégiques dans les domaines de l’énergie, des matières premières, des semi conducteurs, de la santé, du numérique et de la sécurité alimentaire, ainsi que le renforcement des capacités européennes en matière de défense. En l’espace de deux ans, l’Union a été au rendez vous de ces promesses en donnant une impulsion décisive à la politique industrielle européenne le travail législatif s’est mis en marche et a abouti à des textes européens ambitieux ayant pour but de renforcer la production et de prévenir de la sorte les pénuries de semi conducteurs et de médicaments, ainsi que de garantir un approvisionnement sûr, diversifié et durable en matières premières critiques. En parallèle, nous sommes parvenus, dans le sillage des engagements pris lors du sommet, à nous affranchir d’une dépendance pourtant bien ancrée à l’égard des combustibles fossiles russes et avons entrepris de relocaliser une partie de la production de technologies énergétiques propres sur le continent européen. Nous devons désormais, dans le contexte du soutien indéfectible à l’Ukraine, renforcer encore notre autonomie et notre résilience. Cela implique en particulier d’achever rapidement la mise en œuvre de l’agenda de Versailles pour libérer l’Union européenne de toutes ses dépendances, notamment sur le volet capacitaire de défense. Nous devons également progresser très vite sur le thème de la sécurité alimentaire.

Face à un environnement stratégique toujours plus instable, il nous faut nous doter sans délai de tous les outils nécessaires et, surtout, produire, acheter et investir davantage en Européens. Ce changement d’échelle est plus que jamais nécessaire pour fournir à l’Ukraine la profondeur stratégique dont celle ci a impérativement besoin, mais aussi pour renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement de nos armées et préparer l’avenir. Ainsi, il est dans notre intérêt collectif d’envoyer un signal clair et d’assumer une ambition renouvelée pour l’investissement dans les capacités de défense européennes, en mobilisant pour ce faire toutes les ressources européennes à notre portée, y compris l’emprunt, l’emprunt, le recours à la Banque européenne d’investissement (BEI), la mobilisation des intérêts des avoirs russes, dans le respect du cadre juridique que nous avons adopté, ou encore le recours à l’épargne privée. De cela dépendra notre crédibilité face à la Russie en tant qu’alliés de l’Ukraine et vis à vis de nos partenaires de l’Otan. Dans la perspective des échéances à venir, il convient d’expliquer de manière très claire à nos concitoyens le tournant décisif pris par l’Union européenne depuis le déclenchement de la guerre d’agression russe en Ukraine. L’Europe contribue à la sécurité collective et protège les citoyens européens. Disons le clairement, en renforçant les capacités de défense de l’Union européenne, il ne s’agit pas de créer une alternative à l’Otan, c’est tout l’inverse : une Europe qui assume davantage de responsabilités pour sa propre sécurité et qui se donne les moyens de le faire nous rend tous plus forts, plus performants, mais aussi plus crédibles aux yeux de nos partenaires. Le Conseil européen se penchera également sur des sujets clés pour l’avenir de notre continent tels que l’élargissement, avec une discussion sur les éléments présentés par la Commission, le cadre de négociations pour l’Ukraine et la Moldavie et le rapport de progrès sur la Bosnie Herzégovine. Vous le savez, à l’aune du conflit en Ukraine, la France défend la nécessité géopolitique d’une Europe élargie, comme l’a rappelé avec force le Président de la République au printemps dernier lors de la conférence du GlobSec – pour – à Bratislava. Je rappelle également que, dans la perspective de l’élargissement, c’est l’adoption d’un agenda politique clair, notamment à travers l’agenda stratégique, qui nous permettra de définir les réformes opportunes et nécessaires qui garantiront un fonctionnement efficace Le Conseil européen se penchera évidemment sur la situation au Proche Orient, en insistant notamment sur l’urgence à faire appliquer le droit international humanitaire à Gaza, conformément à nos valeurs. Enfin, puisque le sujet des migrations sera également abordé, nous avons affirmé dès 2017 qu’une Europe plus souveraine devait être en mesure de maîtriser ses frontières. À ce titre, l’accord historique sur le pacte sur la migration et l’asile permettra de doter l’Union européenne d’une politique migratoire et d’asile européenne solide, cohérente et efficace. En parallèle, concernant la dimension externe, il nous faut intensifier notre dialogue avec les pays partenaires afin de prévenir les départs irréguliers et d’améliorer la coopération en matière de retour. sont, en quelques mots, les principaux sujets qui seront abordés au Conseil européen de cette semaine. Vous le constatez, ils traduisent au fond une forme de victoire idéologique du logiciel français de souveraineté européenne. Ma conviction est que nous devons à présent poursuivre cette dynamique ambitieuse de réduction des dépendances et de renforcement de la souveraineté en achevant rapidement la mise en œuvre de l’agenda de Versailles, tout en le renforçant. Avec le Président de la République, c’est bien le message que nous porterons au Conseil européen jeudi et vendredi. La parole

Les propos du Président de la République du 26 février, affirmant ne pas exclure l’envoi de troupes au sol en Ukraine, ont surpris nos alliés eux ont pris leurs distances. À cela s’ajoutent de nouvelles tensions avec notre partenaire allemand. Dans ces conditions, il n’est même pas besoin de se demander quel effet a produit au Kremlin cette étrange conception de l’ambiguïté stratégique… Mes chers collègues, le sujet est trop sérieux, trop grave, pour donner lieu à des effets de manche : c’est de la sécurité des Français et de l’Europe qu’il s’agit. Au delà de la forme, la manière d’assurer une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance reste à clarifier. Surtout, pour quoi faire ? Au service de quelle stratégie ? S’il s’agit de dissuader les Russes de se rapprocher de la Transnistrie, alors il faudra y consacrer davantage que des formateurs et des démineurs. Notre commission ne cesse de le répéter : le vrai sujet du soutien à l’Ukraine est la fourniture de munitions. Nous ne sommes pas capables de fournir à ce pays les armes et les munitions dont il a besoin. C’est vrai pour la France, mais malheureusement aussi pour l’Europe. La discrétion La discrétion en la matière des États Unis, qui viennent d’accorder à l’Ukraine un maigre paquet d’aide de 300 millions de dollars, n’est pas rassurante. Cette stratégie est elle même compatible avec l’élargissement de l’Union européenne à l’Ukraine À défaut de pouvoir soutenir l’effort de guerre ukrainien et de donner une signification stratégique à l’élargissement de l’Union, la décision du dernier Conseil européen ressemble à une fuite en avant. Nous faisons des promesses d’adhésion à un pays à qui nous n’avons pas été capables de donner le tiers des munitions que nous lui avons promises. Est ce responsable ? Au Moyen Orient, le conflit israélo palestinien menace toujours d’embraser la région entière. À la sidération du 7 octobre a succédé une impuissance totale de la communauté internationale face à une guerre qui se prolonge et à une situation humanitaire chaque jour plus catastrophique. La France prend sans doute sa part dans la recherche de solutions, mais la capacité d’initiative européenne semble pour le moment bien faible, alors même que les pays européens sont depuis longtemps des bailleurs majeurs du processus de paix au Proche Orient. Certains États membres ont fait des propositions audacieuses, comme l’Espagne et l’Irlande, qui demandent une évaluation, voire une remise en cause de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. La Belgique, que son rôle de présidente du Conseil contraint pourtant à la neutralité, a estimé que la question méritait d’être posée. Comment rapprocher les positions européennes sur ce conflit ? Quelle position la France portera t elle sur ce sujet si sensible à l’occasion du Conseil européen ? Monsieur le ministre, la recomposition violente du monde se poursuit ; on pourrait même soutenir qu’elle s’accélère. Les pays européens doivent jouer tout leur rôle et préserver les intérêts de nos populations – à commencer par leur sécurité mais cela suppose que nous disposions d’une stratégie commune et que nous soyons capables collectivement de défendre des positions fortes et claires. Monsieur le ministre, nous attendons que le Gouvernement agisse en ce sens à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil européen.

à saluer un certain nombre d’initiatives qui ont été prises, en particulier tout dernièrement par la République tchèque, pour approvisionner l’Ukraine en munitions

pour faire monter en puissance la capacité européenne à produire des obus, notamment de 155 millimètres, avec une augmentation de 40 % depuis un an. L’objectif est d’atteindre le plus rapidement possible le million d’obus dans le courant de l’année 2024, puis les deux millions d’obus en capacité de production sur le territoire européen. Le programme et la stratégie présentés le 5 mars par la Commission européenne

et sur les efforts à consentir pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire si importante à Gaza, où la situation est injustifiable

marquer le lancement du semestre européen de 2024. Je rappelle qu’il s’agit là d’un parcours annuel de coordination des politiques économiques et budgétaires nationales, dans lequel s’inscrit

Ils discuteront en particulier de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro préparée par la Commission, d’ores et déjà approuvée par le Conseil. La lecture de ce document me paraît tout à fait instructive, monsieur le ministre, puisque celui ci recommande la mise en d’une politique budgétaire plus restrictive visant à reconstruire des marges de manœuvre budgétaires et à rétablir la viabilité de nos finances publiques. Or la France semble bien loin de cet objectif. objectif. Alors que les prévisions de la Commission anticipent une baisse de 2,8 points du ratio dette sur PIB de la zone euro, lequel atteindrait alors un peu moins de 90 % à la fin de l’année 2024, la France, elle, continue imperturbablement de s’endetter

c’est maintenir un équilibre entre soutenabilité de nos finances publiques et préservation de nos capacités d’investissement. Monsieur le ministre, pouvez vous nous indiquer quelles réformes structurelles permettant de dégager de telles économies seront présentées dans le programme de réformes

Je rappelle, par ailleurs, que la réforme des règles budgétaires européennes qui vient d’être négociée en février 2024 doit entrer en vigueur dans les prochains mois. Certes, la France a réussi, au cours des négociations, à obtenir un assouplissement temporaire pour la période 2025 2027,

que, si le cadre de gouvernance économique révisé s’appliquait aujourd’hui, il se traduirait par une orientation budgétaire plus restrictive que celle qui est actuellement mise œuvre. Ne nous méprenons pas : si la révision des règles budgétaires européennes comporte des incitations à l’investissement public, elle vise principalement à assurer la soutenabilité des finances publiques des États membres. Monsieur le ministre, j’encourage une nouvelle fois le Gouvernement à adopter une position de sérieux budgétaire et à anticiper l’entrée en vigueur du pacte de stabilité et de croissance révisé, en engageant une véritable réduction de notre déficit public.

Vous avez également rappelé que le pacte de stabilité et de croissance a fait l’objet d’une révision, à propos de laquelle la France s’est

le soutien à l’Ukraine, la stratégie européenne de sécurité et de défense, et l’agriculture. Au bout de deux ans, la guerre en Ukraine arrive à un point de bascule où l’unité européenne est mise à l’épreuve. Le chancelier allemand refuse de livrer à l’Ukraine des missiles Taurus à longue portée et, au sein même de sa coalition, certains appellent au gel du conflit quand, de ce côté ci du Rhin, le Président de la République prend l’initiative et envisage même l’envoi de troupes au sol – il a depuis lors nuancé ses propos. Même si le sommet tripartite en format Weimar de vendredi dernier a débouché sur l’annonce d’une coalition de capacité d’artillerie entre Paris, Berlin et Varsovie, il ne suffit pas à résorber les divergences stratégiques de fond qui séparent la France de l’Allemagne et qui sont préoccupantes, à l’heure où le Président Poutine guette les signes de faiblesse de l’Union européenne. La semaine dernière, notre assemblée a confirmé son appui à un soutien durable à l’Ukraine, car elle est convaincue que le prix d’une défaite serait supérieur à celui d’un tel soutien. notre pays peut il valablement tenir longtemps cette ligne alors qu’il n’a aucune marge budgétaire, comme le rapporteur général vient de nous en faire la démonstration Il faut déjà convenir du financement de la nouvelle enveloppe de 5 milliards d’euros que l’Union vient d’accorder à l’Ukraine la Facilité européenne pour la paix. Monsieur le ministre, parviendra t on à mobiliser à cet effet 3 milliards d’euros tirés des revenus des avoirs russes gelés, comme l’espère la France ? En outre, l’Ukraine risque d’avoir encore besoin d’aide d’ici à l’été. Comment financer cette nouvelle tranche ? L’enjeu est de construire une architecture durable de sécurité en Europe, capable de faire face à Vladimir Poutine et peut être, demain, de nous passer d’un éventuel Président Trump. Le soutien à l’industrie de défense européenne nécessite des moyens importants à moyen terme. Cela passe sans doute par l’appui de la Banque européenne d’investissement. Quand celle ci sera t elle autorisée à investir dans ce domaine ? Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour envisager un nouvel emprunt commun. Le Sénat s’en inquiète, déjà soucieux du remboursement de l’emprunt européen levé il y a deux ans pour financer la relance. Monsieur le ministre, pouvez vous nous rassurer ? Un autre sujet d’inquiétude se fait jour en matière de défense

Ces textes ambitieux viennent heurter les compétences des États membres en matière de défense. Or il ne s’agit pas d’une industrie comme une autre. Avec le président Cédric Perrin et les rapporteurs concernés, nous avions déjà alerté à ce sujet la Première ministre, Mme Borne, lors de l’examen par le Parlement européen Jusqu’où le Gouvernement est il prêt à s’en remettre à la Commission pour construire l’Europe de la défense ? Le troisième enjeu de taille du Conseil européen est la question agricole. L’heure de vérité a enfin sonné : la menace qu’un verdissement accéléré de notre agriculture représente pour la souveraineté alimentaire de l’Union est enfin reconnue. Le Sénat n’a cessé de la dénoncer depuis cinq ans, par des résolutions européennes successives ; il se félicite du revirement que représente la révision de la politique agricole commune (PAC), proposée vendredi dernier par la Commission. Enfin, le tabou est brisé. Un « Égalim » européen est même envisagé et nos agriculteurs devraient pouvoir en bénéficier à partir de 2025. En attendant, leurs revenus ne cessent de baisser, leurs contraintes de s’accumuler et les flux d’œufs, de volailles, de sucres et de céréales importés d’Ukraine explosent. Quelles mesures concrètes la France entend elle proposer au Conseil européen pour y remédier ? Ne faut il pas repenser le soutien de l’Union à l’Ukraine, en aidant ce pays à trouver ses marchés habituels ? Monsieur le ministre, il est urgent de secourir nos agriculteurs. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à chaque jalon de la construction européenne, ses défenseurs nous vendent une Europe sociale et une Europe de paix. Il a fallu peu de temps pour que le volet social soit discrédité. Aujourd’hui, après avoir sacrifié les politiques sociales sur l’autel de l’austérité et de la libre concurrence, l’Union européenne prépare la guerre. Si la ligne de front s’est figée, la guerre, elle, ne s’atténue pas pour autant. Cette guerre a jeté 4 millions de personnes sur les routes ukrainiennes, et 6 millions d’autres personnes dans l’exil. Des dizaines de milliers de vies ont été soufflées par les bombes et fauchées par les balles. L’Union européenne doit mettre fin à cette folie et promouvoir des processus de négociation. Nous devons d’urgence élaborer une solution globale de sécurité en Europe et nous affranchir de l’alignement atlantiste, qui ne profite qu’aux États Unis et aux dividendes de guerre. Les coups de menton militaristes du Président de la République, notamment son hypothétique envoi de troupes, sont rejetés en masse par les dirigeants européens.

Monsieur le ministre, je rappelle solennellement que la paix avec la Russie, deuxième puissance nucléaire mondiale, n’est pas une option. Notre jeunesse ne doit pas se préparer à aller au front. La paix est une nécessité existentielle pour les Français, pour les Européens, pour l’humanité. Pour croire en l’avenir, l’humanité doit également avoir confiance dans ses institutions pour relever le défi climatique. La directive dite « Mégacamions » a été adoptée le 12 mars par le Parlement européen. À bien y regarder, le

cinq mètres, soit de véritables immeubles roulants, sans possibilité pour les États membres de s’y opposer. Le désastre écologique est annoncé. Ces véhicules sont neuf fois plus polluants qu’un trajet équivalent le fret ferroviaire. défaut d’investissements et d’une sortie de la logique du tout routier, le fret déraille. Depuis 2000, selon le ministère des transports, le volume transporté a baissé de 43 %. Depuis l’ouverture à la concurrence, en 2007, la situation ne s’est guère améliorée, que l’opérateur historique, Fret SNCF, est en crise. C’est le résultat de ces politiques européennes. Une étude commandée par les entreprises ferroviaires

Les contrats de plan État région et les 900 millions d’euros alloués au fret n’y changeront rien. Un fret sans client, la belle affaire ! À quoi bon avoir inauguré en grande pompe la très pertinente très pertinente ligne Calais Turin si c’est pour la mettre en concurrence déloyale avec ces mastodontes de la route ? Confirmez vous que la France s’opposera, « quoi qu’il en coûte » et jusqu’au bout, à ces mégacamions qui finiront d’anéantir le fret ferroviaire, monsieur comme le ministre Patrice Vergriete, que le report modal est une priorité du Gouvernement ? Sur l’écologie, toujours, sous la pression du patronat, des géants de la finance mondiale, et avec la complicité de la France, la directive sur le

ses investissements et ses produits d’assurance. Autrement dit, la finance verte est définitivement une fumisterie. Nulle conditionnalité des rémunérations exceptionnelles des dirigeants de ces entreprises à l’atteinte d’objectifs climatiques n’ayant été prévue, les actions gratuites vont continuer de se déverser par milliards. La lutte contre la réduction des conséquences des activités humaines sur notre environnement ne peut plus être sacrifiée aux intérêts financiers, le tout

la sénatrice, que cette proposition induirait un report modal inversé, autrement dit une augmentation du transport routier au détriment d’autres modes de mobilité moins carbonés, ce qui serait contraire à notre ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous sommes donc attachés à trouver un compromis plus équilibré entre les enjeux de limitation des émissions du transport routier, de compétitivité économique et de préservation de l’état des infrastructures, et avons proposé que la directive limite la circulation transfrontalière des véhicules dépassant la limite de poids à des trajets inférieurs à 150 kilomètres, ce qui empêcherait la traversée de la France

pour ensuite mettre tous les moyens diplomatiques à sa disposition pour amputer la législation européenne. C’est vrai pour le devoir de vigilance, c’est vrai pour les travailleurs des plateformes,

sans laquelle nous savons qu’un électeur sur deux ne se déplacera pas lors des prochaines élections européennes. J’estime que vous en porterez une part de responsabilité,

ne peut de même que souscrire à la déclaration des ministres des affaires étrangères européens sur la tenue de la prétendue élection présidentielle dans les territoires ukrainiens temporairement occupés en Crimée et dans les quatre oblasts d’Ukraine orientale. Dans ce contexte où le dirigeant russe se sent légitimé à poursuivre son destin impérialiste, le soutien européen à Kiev doit redoubler d’efforts. La France, fortement encouragée par les pays baltes, en était convaincue.

Je pense en particulier à la mise en place d’une véritable industrie de défense mutualisée. Depuis le début de la guerre, 75 % des achats d’équipements militaires sont allés à des firmes non européennes, dont 68 % sont américaines. J’ouvrirai d’ailleurs une parenthèse. Si notre contribution financière à l’Otan est parfois jugée insuffisante outre Atlantique, j’invite nos amis américains à considérer le volet commercial, qui les sert plus que de raison. Si mon groupe approuve la création du fonds d’assistance à l’Ukraine, doté de 5 milliards d’euros, je m’interroge sur la part des achats conjoints européens qui reviendra à l’industrie de défense européenne. Quoi qu’il en soit ou, devrais je dire, quoi qu’il en coûte, mon groupe rejoint la position défendue par la France, la Belgique, l’Estonie ou encore l’Espagne concernant un grand emprunt européen pour financer des investissements dans la sécurité économique et la défense. Le Conseil européen sera également marqué par une autre urgence, celle du drame humanitaire qui se joue depuis octobre dernier dans le territoire de Gaza. Chaque jour, des milliers de civils continuent de payer le prix de la stratégie mortifère du Hamas, qui conduit à la réplique sans réserve de l’armée israélienne. Le RDSE a toujours soutenu la position française : demande d’un cessez le feu immédiat, retour des otages et éradication du Hamas et des colons israéliens violents agissant en Cisjordanie occupée. occupée. Les menaces grandissantes à l’écart des Palestiniens de Rafah nous inquiètent. Une opération militaire d’envergure à la frontière avec l’Égypte conduirait à encore plus de chaos à Gaza.

Tout doit être mis en œuvre pour que l’aide humanitaire parvienne au peuple de Gaza. L’on ne peut pas opposer à l’acheminement de l’aide des arguments techniques, sauf à ce que ces derniers cachent une posture politique de la part du gouvernement israélien. On ne doit pas laisser la famine s’installer à Gaza, au mépris du droit international. Notre devoir est aussi de veiller à l’application des mesures préventives demandées par la Cour internationale de justice

pour alléger les contraintes environnementales dictées par la PAC seront notamment évoqués. Le RDSE salue les propositions qui répondent aux attentes que les agriculteurs français ont exprimées dans la colère durant plusieurs semaines. Enfin, je profite de cette tribune pour saluer les travaux de la Commission et du Parlement sur la régulation des systèmes d’intelligence artificielle (IA). À l’ère de la reconnaissance biométrique à grande échelle, de la propagation des vidéos, de la surveillance de masse et de la notation sociale des citoyens, nous devons nous montrer intransigeants sur ce qui ne peut pas être permis. Monsieur le ministre, la France s’est longtemps opposée à l’IA.

dénoncer les prétendues élections dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, que nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais. Nous avons bon espoir que

Il s’agit généralement du scrutin le moins suivi par nos compatriotes, celui qui souffre du plus fort taux d’abstention de tous nos scrutins. La réforme de 2018, qui a rétabli la circonscription nationale unique, a peut être favorisé une participation un peu plus élevée au scrutin de 2019,

Pourquoi ne pas imaginer spécifiquement pour le scrutin européen, en sus du critère de parité, un critère de répartition géographique des candidats composant une même liste ? En attendant cet éventuel apport au prochain scrutin européen, j’appelle les différentes listes à veiller à la bonne représentation de tous les territoires, notamment de tous les territoires ultramarins, lors de la constitution des listes. Comme lors des Conseils précédents, l’Ukraine occupera certainement l’essentiel des discussions. La guerre entre la Russie et l’Ukraine est en effet entrée dans sa troisième année. Plus les jours passent, et plus il faut nous préparer à voir ce conflit durer des années. Comme l’a rappelé le Premier ministre la semaine dernière lors du débat sur l’accord bilatéral de sécurité entre la France et l’Ukraine, la victoire de l’Ukraine est indispensable. À défaut, il ne pourrait y avoir de sécurité en Europe. Or, en deux ans, nos capacités à soutenir l’Ukraine militairement se sont à peine accrues, et force est de constater que les sanctions économiques prises pour affaiblir l’économie russe et son industrie militaire tardent à produire leurs effets.

Le système dit de Facilité européenne pour la paix, auquel la France a déjà contribué à hauteur de 1,2 milliard d’euros et dont une réforme doit être adoptée lors de ce Conseil européen, permettra t il enfin d’augmenter nos moyens de production, Nous ne pouvons également que constater les multiples contournements des sanctions par la Russie, avec la complicité de pays tiers, comme la Turquie, pourtant membre de l’Otan. L’Inde absorbe maintenant 40 % des exportations russes de pétrole, contre presque rien avant le conflit, et revend sur le marché européen les produits issus de son raffinage. Ces contournements sont documentés et l’on peut les retracer sans difficulté dans les statistiques des pays voisins de la Russie.

ont bondi de presque 3 milliards d’euros, soit une augmentation de plus de 81 % entre 2022 et 2023. La palme revient au Kirghizistan, qui a augmenté ses importations de biens européens de plus de 1 680 Monsieur le ministre, il est temps d’adopter une réglementation plus stricte pour interdire réellement l’utilisation des produits dérivés du pétrole russe et pour soumettre à autorisation les exportations des biens sensibles, surtout vers des pays qui ne servent manifestement que de plateformes de transit pour le contournement des sanctions européennes. Que prévoit l’Union européenne en la matière ? Le sujet sera t il abordé par la France lors de ce Conseil ? De manière générale, il faut mettre fin à toute forme de dépendance économique et commerciale entre la Russie et les pays de l’Union européenne. Telle est la recommandation n° 1 du rapport intitulé

L’une des conséquences de la guerre en Ukraine est la déstabilisation du secteur agricole, qui s’est cristallisée, en ce début d’année, par des manifestations de grande ampleur dans de nombreux pays de l’Union La peur de la concurrence des produits ukrainiens exemptés de droits de douane s’ajoute en effet aux difficultés générées par l’application de la PAC 2023 2027. Le 31 janvier, la Commission européenne proposait un train de mesures temporaires, la prolongation d’un an de la dispense de mise en jachère de 4 % et un mécanisme renforcé de sauvegarde en cas de perturbation des marchés agricoles par des importations de pays hors Union européenne qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences sanitaires ou environnementales. Monsieur le ministre, je sais d’expérience quelles peuvent être les conséquences de la distorsion de concurrence. J’ai vu la production rizicole guyanaise disparaître en quelques années à cause de la réglementation européenne. À quoi bon imposer des normes restrictives à nos agriculteurs si nous acceptons d’importer à moindre coût des produits qui ne respectent pas ces mêmes normes ? Nous ne protégeons alors ni nos consommateurs ni nos agriculteurs. La France fera t elle entendre sa voix pour mettre fin à cette aberration qui dure depuis bien trop longtemps ? J’en viens enfin aux conséquences de l’adoption, par le Conseil européen, de la directive dite RED III, qui concerne le développement des énergies renouvelables. Cette directive prévoit la création de zones d’accélération des énergies renouvelables dans lesquelles le délai de délivrance des permis de construire ne devra pas dépasser douze mois, la création d’une présomption de l’intérêt public majeur des projets d’énergie renouvelable et la création d’un cadre juridique incitatif pour les carburants renouvelables et bien d’autres innovations dans le domaine. Nous avons jusqu’en 2025 pour transposer cette directive en droit interne. Serons nous prêts, monsieur le ministre ? La fâcheuse habitude française à l’inflation bureaucratique qui ralentit toute démarche ne risque t elle pas de contrevenir aux objectifs de cette directive ?

lors des discussions autour de chacun des dispositifs de soutien financier pour l’approvisionnement en équipement militaire de l’Ukraine, la France est toujours le pays qui insiste le plus pour que la préférence européenne soit prise en compte.

ci comprend 117 nouvelles désignations individuelles, ainsi que des mesures sectorielles ciblées sur la production de drones, mais il s’attache aussi à sanctionner les opérateurs logistiques qui organisent les importations illicites de biens vers la Russie.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur les financements de la défense européenne et sur la candidature d’adhésion de la Bosnie Herzégovine à l’Union

Il aura fallu un an et demi pour mettre en œuvre cette ambition et adopter, le 9 octobre dernier, l’instrument nécessaire, le fameux règlement Edirpa Grâce à ce nouveau dispositif, un remboursement partiel sur le budget de l’Union sera accordé aux États membres pour les acquisitions conjointes faisant intervenir un consortium d’au moins trois États. Le

C’est mieux, mais cela paraît encore peu et très éloigné des enjeux auxquels l’Union européenne est aujourd’hui confrontée. Le second volet de cet effort est le renforcement et le développement de nos industries de la défense, y compris nos PME. Je tiens à remettre au cœur de nos débats la taxonomie de l’Union européenne. Nous avons eu l’occasion, il y a quelques semaines, de dénoncer la frilosité bancaire à l’égard des entreprises de la base industrielle et technologique de défense européenne, qui en est la conséquence. Monsieur le ministre, comment comptez vous faire pour intégrer les problématiques de financement du secteur de la défense dans la définition des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG ? Les chefs d’État et de gouvernement devraient apporter leur soutien à un changement des statuts de la Banque européenne d’investissement lui permettant de financer des projets de défense. Pouvez vous nous confirmer que ce sera bien le cas, et nous préciser à la fois les modalités et le volume des crédits espérés ? J’en viens à mon second point, la candidature de la Bosnie Herzégovine. Il a fallu près de six ans et demi entre la demande d’adhésion à l’Union et l’obtention du statut de pays candidat par cet État, qui Pour 83 % des Bosniaques, favorables à cette adhésion, ce sont six ans de rêve européen, six ans de subventions pour mettre en œuvre les réformes clés prescrites, six ans de quête lointaine d’un État de droit, aussi six ans d’illusions, de conférences en sommets, à n’être considérés que marginalement et traités qu’en cas de crise, par exemple la crise migratoire. Ce Ce sont aussi six ans de novlangue bruxelloise, et six ans à consentir à revoir à la baisse la conditionnalité « argent contre réformes » en échange d’une stabilité de façade. Ce sont enfin six ans de sous estimation de la réalité politique des Balkans, justifiée par le lourd héritage des guerres, mais aussi par un méticuleux travail de sape de la Russie et de la Chine. Oui, cette région produit plus d’histoire qu’elle n’en peut consommer, pour reprendre les propos attribués à Churchill. Le système politique bosniaque est complexe, hérité des accords de paix de Dayton, parfois synonyme de clientélisme et de captation d’État. Ajoutez à cela l’affaiblissement du modèle européen au sein de l’opinion publique

dans la région ? Après les élections européennes de juin, la réforme des traités sera t elle mise sur la table pour qu’enfin la gouvernance européenne soit repensée et son fonctionnement renforcé ? Ce dernier point est un préalable indispensable à tout élargissement.

attachés à une approche fondée sur les mérites propres de chaque candidat. Il est essentiel que le pays mette en œuvre les réformes nécessaires. La crédibilité du processus d’adhésion en dépend. Certes, c’est un

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’ordre du jour du Conseil européen des 21 et 22 mars est de nouveau dominé par des sujets lourds correspondant à de forts enjeux géopolitiques : la situation en Ukraine et celle, tout aussi tragique, au Moyen Orient. Par manque de temps, c’est la seule Ukraine qui sera l’objet de mon intervention. De toute De toute évidence, l’évolution du conflit ukrainien exige que les dirigeants européens se parlent et s’efforcent de définir sur le sujet une ligne claire pour une action commune efficace. Cette réunion devrait fournir une nouvelle occasion Dans cette perspective, il est désolant que le Président de la République ait brouillé les cartes, le 26 février dernier, par des propos inconsidérés, qui ont déconcerté aussi bien les citoyens français que la plupart de nos partenaires européens. Quoi que l’on pense au fond de la position personnelle qu’il a alors exprimée, il faut d’abord déplorer qu’il l’ait fait sans aucune concertation préalable avec le Parlement et les principales forces politiques du pays, la saisine du Parlement venant. Cela est d’autant plus condamnable qu’il est clair que cette sortie était motivée tout autant par des préoccupations de politique intérieure que par un réel souci de positionnement stratégique de la France. Dans son entretien télévisé du 14 mars sur TF1 et France 2, le Président de la République a tenté de s’expliquer auprès des citoyens français. C’est peu dire qu’il n’a guère été compris et que les téléspectateurs sont sortis de ce spectacle plus consternés et effrayés que convaincus et rassurés. Il s’agit maintenant de restaurer la confiance altérée avec nos principaux partenaires européens, au premier chef desquels l’Allemagne, avec qui nos relations bilatérales n’ont pas été aussi tendues depuis très longtemps. C’était l’objet du voyage du Président de la République à Berlin, vendredi dernier, et ce sera de nouveau l’objet des discussions qui auront lieu à Bruxelles cette semaine, dans le cadre du Conseil européen. Dans le contexte actuel de confrontation exacerbée avec le régime russe de Poutine et d’une possible défection des États Unis dans quelques mois, la division des Européens est inconcevable. L’heure n’est pas à la forfanterie et aux discours martiaux ; elle est à l’action concrète, collective et proportionnée pour soutenir l’Ukraine. Les efforts déployés jusqu’à présent par l’Union européenne sur tous les plans sont considérables et se chiffrent en dizaines de milliards d’euros. Mais, sur le plan strictement militaire, notamment pour ce qui concerne les armes et les munitions, ils sont encore insuffisants. L’un des enjeux de la réunion du Conseil européen sera donc de mobiliser de toute urgence les moyens nécessaires pour empêcher que le front ukrainien ne cède. Spéculer à ce stade sur ce que pourraient éventuellement être les degrés suivants d’une escalade n’est utile ni pour le bien de l’Ukraine ni pour les intérêts européens. Au risque de me répéter, je ne considère pas non plus que la perspective d’une adhésion future de l’Ukraine à l’Union européenne contribue en quoi que ce soit à la résolution du conflit en cours. Elle ne peut, au contraire, que frustrer l’Ukraine, en lui donnant de faux espoirs, et provoquer la Russie en justifiant son discours sur une prétendue menace occidentale à ses frontières. L’Ukraine ne remplit quasiment aucun des critères requis pour une telle adhésion – nous le savons bien. En effet, il s’agit d’un pays dont l’appareil productif n’est certainement pas en état de permettre une intégration harmonieuse dans l’union douanière et le marché unique européens. L’ouverture sans restriction du marché de l’Union européenne aux produits agricoles ukrainiens dans le cadre des mesures autonomes de libéralisation a déjà sérieusement perturbé les marchés européens des céréales, de la volaille, des œufs et du sucre. Selon une évaluation du secrétariat général du Conseil, si l’Ukraine devenait membre de l’Union européenne, elle pourrait prétendre, suivant les critères en vigueur, à 96 milliards d’euros de fonds de la PAC, ce qui entraînerait une réduction d’environ 20 % des subventions agricoles accordées aux États membres actuels. Le vice ministre ukrainien de l’économie a lui même reconnu que cela entraînerait la fin de la PAC telle que nous la connaissons aujourd’hui. Je voudrais donc conclure mon intervention par un appel à la plus grande prudence. Cessons d’agiter des idées extravagantes lorsque nous ne sommes pas forcément capables d’en assumer toutes les conséquences.

que le Président de la République, le 26 février dernier, était mû par des motifs de politique intérieure. Eh oui ! Mais alors, comment expliquez vous que vingt six chefs d’État et de gouvernement aient répondu à son invitation alors qu’une grande majorité d’entre eux ne sont pas sur la même ligne politique que lui ? semblez vouloir dire – que le Président de la République a eu tort de n’exclure aucune option. Mais alors, je vous le demande, monsieur le sénateur : quelles sont les options qu’il eût fallu exclure ? relation de confiance avec l’Allemagne est au plus bas. Mais alors, comment qualifier les relations très intenses qui se sont nouées, ou en tout cas qui

l’accueil que j’ai réservé à ma propre homologue à Paris, la semaine dernière, la participation à notre dernier conseil des ministres de la ministre de l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne, ou bien encore, au niveau parlementaire, le colloque célébrant les cinq ans de l’Assemblée parlementaire franco allemande pendant lequel il a été fait état de

le sommet de jeudi et de vendredi constituera le dernier Conseil européen « ordinaire » avant les élections des 6 au 9 juin, qui qui pourraient aboutir – nous le savons tous – à une poussée des populistes au Parlement européen. Dans ce contexte, le Conseil européen, qui définit les grands axes de la politique de l’Union européenne, doit poursuivre son action au service de tous les Européens pour la paix, la sécurité et la prospérité de notre continent. Comme l’a rappelé le Président de la République, la situation évolue en Ukraine à grande vitesse et pas dans le bon sens. C’est pourquoi l’adoption par le Sénat et l’Assemblée nationale de l’accord de sécurité entre la France et l’Ukraine, la semaine dernière, a été un acte fondamental. C’est pourquoi, aussi, l’action de l’Europe est indispensable. La passivité n’est plus de mise. Nous ne pouvons pas nous contenter de ne pas agir. Ces deux dernières années, l’Union européenne et les États européens ont fourni un soutien financier et militaire

entre le Président de la République française, le chancelier allemand et le Premier ministre polonais a permis de réaffirmer un soutien indéfectible De même, les déclarations appelant à une industrie européenne de la défense capable de produire enfin à grande échelle vont dans le bon sens. Je salue ces efforts, mais l’évolution de la situation en appelle d’autres, notre destin étant intrinsèquement lié à celui de l’Ukraine. Dans cette perspective, monsieur le ministre, pouvez vous nous préciser si le sujet du nouvel emprunt européen évoqué pour aider l’Ukraine sera en discussion à partir de jeudi prochain ? Pouvez vous également nous en expliquer les contours ?

comment la France compte t elle faire la différence pour enfin œuvrer activement à la mise en place d’une défense européenne ?

Je sais que le Gouvernement est très engagé et à l’écoute sur ce sujet. L’Europe semble avoir entendu la détresse du monde agricole, non seulement français, mais aussi européen, puisque la Commission a proposé, vendredi dernier, une évolution des règles de la PAC.

Dans ce contexte, monsieur le ministre, quelles mesures allez vous porter en matière agricole durant ce Conseil ? La simplification des normes et des règles administratives est cohérente, mais de certaines règles de la PAC et de la révision de la stratégie « de la ferme à la fourchette

le ministre délégué. Monsieur le sénateur, l’idée d’un emprunt européen a été initialement portée par la Première ministre estonienne.

l’idée d’explorer cette voie pour répondre aux besoins importants nécessaires à l’émergence ou au réveil de notre base industrielle et technologique de défense.

Madame la présidente, monsieur le ministre,

Mon intervention concernera l’Ukraine et sa demande d’adhésion à l’Union européenne. Je crois, en effet, qu’il faut bien faire la distinction entre le soutien que nous devons lui

En effet, monsieur le ministre, le parcours d’adhésion de l’Ukraine doit respecter les critères de Copenhague. L’état de guerre entre l’Ukraine et la Russie ne doit pas nous

soit considérée comme un candidat sérieux, doit encore faire face à des défis majeurs – il faut être lucide sur ce point – comme la corruption ou l’influence persistante des oligarques. D’ailleurs, la présidente de la Commission européenne la présidente de la Commission européenne semble avoir pris la mesure des difficultés que pouvait engendrer une adhésion trop rapide de l’Ukraine à l’Union. En effet, elle a récemment indiqué que la feuille de route politique des négociations serait prête non pas avant les élections européennes, mais plutôt

son processus d’adhésion à l’Union européenne, afin de satisfaire aux obligations requises pour cela. Ce postulat illustre bien qu’il reste encore du chemin à parcourir pour que l’Ukraine concrétise son adhésion à l’Union européenne.

pour l’Ukraine, dont 17 milliards d’euros de subventions et 38 milliards d’euros de prêts. Cette aide, pleinement justifiée, comporte notamment le plan Ukraine par lequel le gouvernement ukrainien présentera ses intentions pour le redressement, la construction et la modernisation Au titre de l’investissement pour l’Ukraine, l’Union européenne fournira un soutien sous la forme de garanties budgétaires et d’une combinaison de subventions et de prêts d’institutions publiques et privées.

absolument indispensable – à ce que le processus d’adhésion reste fidèle au principe sur lequel il est fondé, c’est à dire les mérites propres du pays candidat. L’Ukraine a engagé un certain nombre de réformes qui ont conduit les chefs d’État et de gouvernement à décider l’ouverture des

d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, nous avons élargi avant d’approfondir. Je ne suis pas du tout pessimiste sur la question de l’unité et de la souveraineté, mais je pense que cela doit aller de pair avec une réforme institutionnelle forte. C’est seulement dans un deuxième temps

présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les 5 milliards d’euros pour l’Ukraine sont une bonne nouvelle. Face au retrait du Congrès américain et face au risque d’une nouvelle offensive russe, cette enveloppe est un soulagement. monsieur le ministre, que de blocages pour en arriver là ! L’Allemagne préférait privilégier les aides bilatérales, la France mettait le comme condition : était il bien raisonnable de bloquer les négociations pour cela ? Il a quand même fallu huit mois pour aboutir

me semble que la liberté et la résistance de l’Ukraine nous obligent à des garanties plus durables. Il faut en effet utiliser les milliards d’euros générés par les avoirs russes gelés.

Pour juguler l’impérialisme de la Russie de Poutine, pour raffermir le droit international, pour que la sécurité et la paix ne soient pas subordonnées à l’hypothèque électorale étasunienne, il est temps de faire mieux et d’agir en d’agir en Européens en mettant fin à cette diplomatie menée en solitaire qui déstabilise nos concitoyens, nos alliés et donc le soutien à l’Ukraine. Ne croyons pas non plus que la voie de la paix soit celle des exhortations à de prétendues négociations immédiates avec l’envahisseur russe, pseudo négociations qui mettraient dans un grand chaudron les revendications d’expansion russe sur les territoires russophones, ici et là, une neutralité imposée pour ce qui resterait de l’Ukraine, la question de l’Otan et celle de l’Union européenne. Je crois que de telles exhortations sont, de fait, un message d’incitation à l’escalade guerrière, puisqu’elles admettent que des territoires trop faibles pour se défendre peuvent être obtenus par la force. Pour que ne faiblisse pas le soutien des Français à l’Ukraine, ne laissons pas se propager le sentiment d’un deux poids, deux mesures, s’agissant de la détermination de notre pays, entre Kiev et Gaza. Depuis l’horrible attaque terroriste du Hamas et la détention des otages,

rarement égalée, ainsi que par les ravages de la faim et des privations. Aujourd’hui, face à ce que le Haut Représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, qualifie de situation d’insécurité alimentaire aiguë pour les Gazaouis face à la famine utilisée comme arme de guerre, le Conseil européen doit clairement changer de registre à l’égard du gouvernement d’Israël et exiger le cessez le feu et l’accès complet à l’aide humanitaire. Pour cela,

L’Union européenne verserait donc inconditionnellement une telle somme à un régime répressif qui compte quand même plus de 60 000 prisonniers politiques et où la corruption est généralisée. Quel cynisme de servir de cette façon de banque aux régimes dictatoriaux ! Notre pays soutient il sans réticence la logique de cet accord consternant ? Nous nous interrogeons aussi sur le rôle contre productif qu’a joué la France dans deux chantiers législatifs européens qui sont arrivés à leur terme. Je déplore ainsi que la France ait œuvré pour amputer toute ambition à la directive sur le devoir de vigilance des entreprises et qu’elle se soit évertuée, seule contre tous, à soutenir les plateformes contre leurs travailleurs précaires.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les règles budgétaires de l’Union européenne s’appliquent de nouveau depuis janvier 2024 après avoir été suspendues en 2020. Un nombre important d’États membres, dont la France, risquent de faire l’objet d’une procédure pour déficit excessif. L’exécutif communautaire a pourtant bien perçu l’urgence qu’il y a à assouplir les normes en vigueur : l’accord obtenu en février dernier sur une réforme du pacte fiscal européen est ainsi censé attribuer plus de flexibilité aux États membres.

aux gouvernements nationaux d’intervenir dans leurs économies. Les États membres de l’Union ont franchi un pas supplémentaire et opéré un changement de paradigme économique, en acceptant d’emprunter en commun pour financer le plan de relance européen.

L’application de critères chiffrés uniformes – ceux de la dette publique et du déficit – paraît dès lors absurde, contre productive d’un point de vue économique et dangereuse politiquement. Un retour en arrière, vers une forme de conservatisme budgétaire, est impensable au moment où les États membres doivent plus que jamais investir dans la transition écologique, l’éducation, l’industrie verte et la défense.

Une véritable refonte du cadre et de la surveillance budgétaires, qui inclurait les investissements prioritaires européens et permettrait de tenir compte de la conjoncture économique de chaque pays, nous paraît aujourd’hui indispensable. Pouvons nous réellement nous contenter des mesures cosmétiques de la réforme du pacte de stabilité et de croissance ?

à l’unanimité et qui a donc supposé des discussions longues et particulièrement serrées avec nos partenaires, au premier rang desquels figurait notre voisin allemand. Je crois que cette évolution ne pourra pas nuire.

je le revendique, je le confirme, est un concept que la France a progressivement fait entrer dans la grammaire européenne. Atteindre cet objectif supposera évidemment la mobilisation de l’épargne et de financements privés, mais aussi de ressources publiques. Cela doit nous amener à réfléchir à la manière dont nous pourrions – comme nous l’avons fait face à d’autres impératifs ou à d’autres urgences, en 2020 par exemple

Alors que le ramadan a débuté le 11 mars courant, sans que les négociations visant à obtenir une pause humanitaire immédiate aient pu aboutir, 1,1 million de Gazaouis se retrouvent donc confrontés à la faim, dans une situation catastrophique, proche de la famine selon l’ONU.

Un premier navire, chargé de 200 tonnes de nourriture, représentant environ 300 000 repas, est finalement arrivé à bon port vendredi dernier et sa cargaison a pu être déchargée. L’envoi d’un second navire a été annoncé dans la foulée. étant, la taille des bateaux et, donc, le volume de l’aide fournie restent limités face à l’ampleur des besoins, d’autant qu’il n’y a pas de port pour décharger la marchandise à Gaza. La donne pourrait cependant changer prochainement, car les États Unis ont prévu la création d’un port flottant dont la construction devrait prendre soixante jours.

Nous avons constaté que plusieurs de ces pays étaient parvenus à prendre des mesures pour se conformer aux critères de Copenhague, en vue de leur adhésion. Ces critères exigent notamment des pays candidats que ceux ci respectent les principes démocratiques, l’État de droit et les droits de l’homme. ces standards constitue une étape préliminaire fondamentale à l’ouverture des négociations d’adhésion. Toutefois, il convient de rester attentif et de ne pas confondre vitesse et précipitation.

qui concerne les contributions financières des États, le budget de l’Union et la répartition des aides européennes, donc vigilance sur les conséquences économiques qui en résulteront. Notre pays et l’Allemagne sont contributeurs nets de l’Union

de la France n’est absolument pas d’aller dans le sens d’une suspension de cet accord. Au contraire, l’Union européenne, même au delà de ses frontières, doit rester particulièrement attentive à la situation en Israël et à Gaza.

nous voyons bien que l’Europe est désirée, et ce bien au delà de nos frontières. Soyons conscients de la chance que nous avons, soyons fiers de l’Europe et soyons fiers d’être Européens ! La parole est à M. le ministre délégué.

de la France sur le fait – c’est d’ailleurs un principe que nous réaffirmons très régulièrement – qu’il ne peut pas y avoir d’élargissement réussi si, en parallèle, il n’y a pas une triple réforme de l’Union européenne. Tout d’abord, une réforme des politiques parce que la politique agricole commune et la politique de cohésion doivent permettre d’accueillir les pays candidats, sans déstabiliser

niché au cœur des Balkans occidentaux, dont la plupart des voisins sont engagés dans un processus d’adhésion et qui, le moment venu, basculera sans doute

commune appelant à un cessez le feu durable, à l’acheminement de l’aide humanitaire et à la dénonciation de l’attentat terroriste du Hamas, ce qui permettrait de souder

avec en toile de fond les dernières déclarations du Président de la République, qui n’ont pas manqué de déconcerter nos alliés et d’inquiéter les Français. Le sujet de mon intervention ne sera pas original, mais il ne se passe pas un seul jour sans que nous soyons interpellés par nos concitoyens préoccupés par le changement de discours du Président de la République. dernier affirmait voilà quelques mois encore qu’il ne fallait pas humilier la Russie, il n’exclut plus aujourd’hui l’envoi de troupes sur le front. Bruno Retailleau a rappelé la semaine dernière la position claire et sans ambiguïté de notre groupe tout faire pour que la Russie ne remporte pas ce conflit ; ne rien faire qui nous entraîne dans une guerre dont nous ne voulons pas. Nous jugeons également que la promesse d’une adhésion rapide de l’Ukraine à l’Union serait prématurée, car cela entraînerait des conséquences sociales et économiques délétères pour la France, à commencer par une baisse du budget de la PAC du fait de l’importance de la surface agricole ukrainienne. Nous voyons déjà aujourd’hui les conséquences de l’ouverture sans contrôle du marché européen aux produits agricoles ukrainiens : des prix cassés et nos agriculteurs en grande difficulté face à une concurrence déloyale, qui produit sans avoir à respecter les mêmes normes que nous. Je profite de l’occasion, monsieur le ministre, pour réitérer la question que j’ai posée ici même il y a quinze jours à votre gouvernement et à laquelle je n’ai pas eu de réponse : êtes vous ou non favorable aux clauses de sauvegarde pour limiter les importations de céréales ukrainiennes et protéger ainsi nos producteurs ? Le Conseil européen se penchera aussi sur la politique agricole commune. Vendredi dernier, la Commission européenne a enfin accepté de briser le tabou de la réouverture de la PAC, en remettant pour la première fois en cause son architecture verte. La suppression de l’obligation de jachères, l’assouplissement de rotation des cultures et de couverture des sols en hiver, ou encore la réduction des contrôles sont autant de mesures qui vont dans le bon sens. Toutefois, que de temps perdu ! Toutes ces préconisations figuraient déjà dans de multiples résolutions et rapports publiés par le Sénat depuis 2017. Reste désormais à savoir comment ces propositions seront appliquées. Nous appelons à une grande vigilance face au risque de renationalisation de la PAC et à la manière dont la France se saisira de cette nouvelle flexibilité. Ce sujet ne doit pas se cantonner à un simple discours de campagne pour les élections Dans le domaine de la santé, je me réjouis qu’un compromis ait été trouvé à Bruxelles sur l’espace européen des données de santé. Il est essentiel de favoriser la recherche sur le territoire européen, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel de nos concitoyens. été conclu reprend d’ailleurs l’une des dispositions que nous proposions, à savoir la possibilité pour les patients de s’opposer au traitement de leurs données de santé à des fins de recherche. données de santé, nous demandions également que les données de santé électroniques et les services associés soient hébergés sur le territoire de l’Union européenne, par une entreprise européenne. Aussi, je regrette que le gouvernement français s’obstine à vouloir confier à Microsoft l’hébergement des données de santé des Français…

que vous nous indiquiez comment vous entendez la transposer en droit français. Pour conclure, mes chers collègues, j’insiste sur le fait que nous attendons de ce sommet européen des mesures fortes de soutien à l’Ukraine sans pour autant tomber dans le bellicisme ; nous attendons des mesures puissantes pour sauver nos agriculteurs ; nous attendons de la France plus de constance et de clarté pour continuer de tenir son rang

nous sommes d’ores et déjà victimes de l’agressivité de Vladimir Poutine. Qui a fait flamber les prix du gaz pour nos concitoyens ? C’est Vladimir Poutine ! Qui inonde les marchés mondiaux de céréales à prix cassés, ce qui fragilise nos agriculteurs ? C’est Vladimir Poutine

Qui a, encore aujourd’hui, diffusé une fausse nouvelle sur l’envoi présumé de troupes françaises en Russie ? Ce sont les services de renseignement russes ! Bref, nous sommes soumis à une agressivité très forte